: La parole est à M. François Bonhomme. Cet amendement vise à interdire aux membres du Gouvernement d'adresser à l'administration des impôts des instructions dans des affaires individuelles, dans le cadre de la délivrance de l'attestation fiscale prévue par le présent projet de loi. En effet, tel que le prévoit l'article 30 du code de procédure pénale s'agissant des rapports du garde des sceaux avec les magistrats du ministère public, il paraît nécessaire de prévenir l'ingérence des membres du Gouvernement dans cette procédure, qui relève strictement de l'administration fiscale.

dans le cadre de la délivrance de l'attestation fiscale que la loi exigera de tout élu au Parlement. Cela devrait aller sans dire. Nous pensons que cela va mieux en le disant

à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a posé, l'année dernière, les premiers éléments d'une protection des lanceurs d'alerte dans le secteur public. En l'état actuel des choses, tout fonctionnaire ou agent du public ayant pris connaissance d'un crime ou d'un délit au sein de la collectivité ou de l'établissement public dans lequel il travaille est tenu d'en informer le procureur de la République. C'est essentiel, mais c'est insuffisant, puisque la loi ne précise aucune obligation à l'exercice de ce devoir. En effet, aujourd'hui, aucune sanction ne peut être prise en cas de manquement. Notre amendement a pour objet d'y remédier. Cet amendement est aussi un appel en direction du Gouvernement, avec pour objectifs, premièrement, de mieux définir dans quel cadre et sous quel régime de sanction pénale un fonctionnaire a le devoir et l'obligation de faire part au procureur de la République de tout crime ou délit dont il sera témoin et, deuxièmement, de continuer à légiférer à ce sujet, notamment parce que la déontologie actuelle ne concerne que les délits et les crimes, ce qui n'inclut pas, par exemple, les risques sérieux pour la santé publique ou même les risques environnementaux. Renforcer l'obligation pour les fonctionnaires et agents d'informer le procureur de la République lorsqu'ils ont pris connaissance d'un délit ou d'un crime, c'est d'abord mieux protéger les lanceurs d'alerte du secteur public. C'est aussi accroître la confiance de nos concitoyens dans l'action publique.

Gouvernement ? Cet amendement prévoit une sanction pénale en cas de non-respect des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale. à l'obligation prévue par le second alinéa de l'article 40 peut exposer un agent public à des poursuites disciplinaires, voire pénales, en cas de complicité, sur le fondement de l'article 121-7 du code pénal, ou de non-dénonciation de crimes, sur le fondement de l'article 434-1 du même code. En outre, sanctionner pénalement les fonctionnaires qui ne dénonceraient pas des comportements délictuels pose, selon nous, deux types de difficultés. D'une part, cela pourrait inciter les fonctionnaires à ne prendre strictement aucun risque, donc à dénoncer massivement dès lors qu'un doute naîtrait dans leur esprit. D'autre part, il serait difficile de démontrer que la personne ne pouvait pas ignorer le caractère frauduleux du comportement qu'elle aurait dû dénoncer. Pour ces raisons, nous émettons un avis défavorable

Saisie par le président de l'Assemblée nationale, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP, s'est intéressée à son tour aux clubs parlementaires en 2016. Elle a souligné la grande hétérogénéité de leurs statuts et l'absence d'encadrement juridique. Nous proposons de compléter la loi de 2013 afin de définir les clubs et d'encadrer leur fonctionnement. En plus de les contraindre à une forme associative, notre ces instances de rencontres ne peuvent utiliser le terme de « parlementaire » ou « sénatorial » dans leur dénomination, ne peuvent utiliser le logo du Sénat ou de l'Assemblée nationale, nationale, ne peuvent utiliser le terme de « parlementaire » ou « sénatorial » dans l'organisation de colloques, manifestations, réunions ou dans les documents produits. Le non-respect de ces dispositions, après injonction de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique restée sans effet dans un délai d'un mois, est passible d'une amende de 15 000 euros.

des règles qui relèvent du fonctionnement interne de nos assemblées. Il se trouve que le comité de déontologie de notre assemblée s'est déjà prononcé sur ces règles. Mon cher collègue, vous avez tout à fait raison sur le fond, mais votre amendement n'est pas le bon vecteur. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir le retirer. Quel est

On y apprend que 75,5 % des inspecteurs généraux des finances ont pantouflé- 34 % de façon durable.

des anciens élèves de l'ENA ont pratiqué cette technique sportive de promotion

de trois ans, renouvelable une fois, contre dix ans actuellement. Dans le même temps, il vise à assurer aux magistrats siégeant à la commission de déontologie de la fonction publique, en charge notamment de donner un avis sur de tels cas de mobilité, une majorité de sièges par rapport aux personnalités qualifiées et aux représentants des administrations. De la sorte, les contrôles existants à l'occasion du passage d'un fonctionnaire du secteur public au secteur privé seraient doublement renforcés.

Notre souci est de rendre plus efficace le contrôle de compatibilité qui affiche aujourd'hui certaines lacunes. Si les détenteurs d'un mandat électif, les animateurs de notre vie politique, se doivent d'être exemplaires, les plus hauts décisionnaires de l'appareil étatique, étatique, tels que les hauts fonctionnaires, doivent également l'être. Il est assez scandaleux de constater que de plus en plus de diplômés de l'ENA ou de l'École polytechnique, pour ne citer que celles-là, pantouflent dans les entreprises sans même avoir respecté leur engagement de dix ans au service de l'État. Nous nous devons de lutter contre ce qui peut s'apparenter à une forme blanche de corruption. Le pantouflage pose de sérieux problèmes éthiques et déontologiques liés au mélange des sphères privée et publique

d'assortir le non-respect de l'engagement de dix ans au service de l'État pour ces hauts fonctionnaires de la radiation de la qualité de fonctionnaire, ainsi que du remboursement d'une partie des frais de scolarité. Quel est l'avis de la commission sur ces différents amendements

la vie politique ne traite aucune question de fond. Elle se borne à recevoir des déclarations d'intérêts et de patrimoine et à vérifier qu'il n'y a pas eu d'enrichissement

au-delà duquel la commission de déontologie n'a plus à examiner la compatibilité entre l'activité du fonctionnaire dans le secteur privé et son activité antérieure dans l'administration. La commission a émis

même temps. Il ne paraît pas possible de définir dans la loi un plafond des effectifs des fonctionnaires mis en disponibilité. En effet, les disponibilités varient d'un corps à l'autre et ne sont pas toutes prises pour réaliser une mobilité vers le secteur privé. Elles peuvent, par exemple, être utilisées par des fonctionnaires

fins lucratives d'un réseau ou d'une clientèle constituée dans le cadre de l'exercice et pour l'objet d'une mission de service public, en introduisant un délai de trois ans pendant lequel un ancien fonctionnaire ne peut exercer une activité de conseil liée à ses anciennes missions de service public. Cette mesure limite provisoirement la mobilité des anciens fonctionnaires vers le secteur privé, permettant de s'assurer de leur plein dévouement à leur mission de service public et de restaurer ainsi la confiance des citoyens dans l'action publique.

publics en disponibilité, et ayant exercé des fonctions pour le compte d'une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil, d'occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l'exercice de prérogatives de puissance publique dans un même secteur d'activité, pendant un délai de trois ans.

l'avis du Gouvernement ? pas me répéter indéfiniment, mais je crois que cela vaut pour un certain nombre d'amendements.

Cet amendement a pour objet de limiter la possibilité pour les anciens fonctionnaires ou agents publics de devenir des représentants d'intérêts auprès ou pour le compte d'une personne morale de droit public dont ils auraient fait partie. Le délai de carence de trois ans introduit dans cet amendement permet de prévenir les situations potentielles conduisant à des prises illégales d'intérêts au sens de l'article L. 432-12 du code pénal et de rétablir ainsi la confiance des citoyens dans l'action publique. Ce dispositif n'interdit pas l'exercice par l'ancien fonctionnaire ou agent public de la fonction de représentant d'intérêts, mais lui impose simplement un délai de trois ans pour le faire auprès de son ancien employeur.

le Gouvernement présente un texte que les parlementaires sont obligés de se plier à sa logique. Exactement ! C'est notre liberté

Monsieur Retailleau, je n'ai ni le désir ni le pouvoir de restreindre la liberté du Parlement, soyez-en sûr, et je respecte absolument tous les amendements qui peuvent être déposés. Je fais simplement part d'une réticence d'ordre juridique, en soulignant que, au regard des dispositions initiales du projet de loi, celles que vous évoquez sur la fonction publique, indépendamment de leur pertinence et de leur légitimité,

le Gouvernement a éprouvé le besoin de faire examiner par le Parlement des dispositions concernant les parlementaires dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions,

sur la déontologie des parlementaires et, à la marge, des membres du Gouvernement et des exécutifs locaux, présente une lacune évidente : aucune mesure ne concerne la haute fonction publique. Pourtant, un phénomène ne cesse d'être constaté en son sein : le « pantouflage » pose de sérieux problèmes éthiques et déontologiques liés au mélange des sphères privées et publiques, et des sphères de l'intérêt général et des intérêts particuliers ou de grandes entreprises. Il est évidemment source de situations de conflits d'intérêts. C'est pourquoi nous proposons que le non-respect de l'engagement à servir l'État pour une durée minimum de dix ans soit assorti de la radiation de la qualité de fonctionnaire, ainsi que du remboursement d'une partie des frais de scolarité.

Pour moraliser l'action publique, il convient parfois- hélas ! -de mettre en oeuvre des dispositions très pragmatiques. Certains hauts fonctionnaires attirés par l'appât du gain réfléchiraient davantage

le rapport dont nous venons d'adopter le principe, avant de prendre de telles dispositions ? J'observe d'ailleurs que celles-ci présentent un caractère discriminatoire.

font une partie de leur vie professionnelle ailleurs que dans l'administration. Pourquoi devrions-nous adopter un amendement qui réserverait les sanctions à une catégorie seulement de fonctionnaires,

à celui dont dispose l'administration fiscale, sur le fondement du livre des procédures fiscales. Cet amendement a pour objet d'adapter ce droit de communication aux besoins réels de la Haute Autorité pour l'exercice de ses missions.

Ensuite, le présent amendement vise à doter la Haute Autorité d'un droit de communication auprès des établissements bancaires et des entreprises d'assurance vie, c'est-à-dire des tiers détenant l'essentiel des informations utiles à la Haute Autorité. Ces droits de communication complètent l'enrichissement des moyens d'enquête de la Haute Autorité, qui disposera prochainement d'un accès direct à plusieurs fichiers de l'administration fiscale, lesquels contiennent un grand nombre d'informations utiles à

la BNDP, la base nationale des données patrimoniales, et de PATRIM, qui recense les prix de cession des biens immobiliers. Enfin, par cohérence, il est proposé que l'administration fiscale n'exerce plus pour le compte de la Haute Autorité son droit de communication pour obtenir les informations que cette dernière pourra désormais recueillir directement. En réalité, il s'agit de donner à la HATVP des pouvoirs importants, mais qui ne sont pas équivalents à ceux d'un parquet. Autrement dit, cet amendement tend à lui conférer une augmentation raisonnable de ses compétences et une augmentation raisonnée de ses pouvoirs. Elle pourra faire finances publiques, la DGFiP, faisait jusqu'alors pour son propre compte. Nous pensons que nous respectons ainsi la logique de la mission de la Haute

par l'administration fiscale, il n'est pas rare que cette dernière ait alors la puce à l'oreille et se mette à procéder à ses propres investigations.

d'atteindre un régime de croisière, demande directement ces informations à ceux qui les détiennent, sans avoir besoin de dévoiler à l'administration fiscale qu'elle s'intéresse particulièrement

que par le biais de la suppression de ce que nous nommons les « emplois familiaux ». Selon nous, la crise de confiance dans l'action publique ne sera pas résolue par l'interdiction des seuls emplois familiaux. Le sujet est bien plus large ; la difficulté est bien plus profonde : il s'agit en réalité d'une crise des institutions de la V République. L'interdiction des emplois familiaux n'apportera pas de solution au réel problème qu'est l'absence de cadre légal de la profession des collaborateurs parlementaires. L'absence d'un statut professionnel des collaboratrices et collaborateurs parlementaires comprenant une fiche de poste, précisant les missions, les qualifications et le niveau de rémunération laisse la porte le niveau de rémunération laisse la porte ouverte aux potentielles dérives, comme la rémunération par les lobbys de certains collaborateurs ou les emplois fictifs. telle situation met à mal l'image de l'ensemble des parlementaires quant à l'usage de l'argent public mis à leur disposition, c'est aussi l'image des collaborateurs qui nous accompagnent au quotidien qui est écornée. Pour y remédier, nous proposons d'étendre les dispositions du texte aux emplois de collaborateur parlementaire, de collaborateur de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, de collaborateur de ministre et de collaborateur d'élu local. Cet amendement a donc pour objet de modifier l'intitulé du titre III du projet de loi, pour répondre à l'exigence de transparence et de rétablissement de la confiance dans l'action publique.

Cet amendement a donc pour objet de modifier l'intitulé du titre III du projet de loi, pour répondre à l'exigence de transparence et de rétablissement de la confiance dans l'action publique. La parole est

dans l'intérêt de ces derniers, mais aussi des employeurs que nous sommes. Elles ne remettent en aucun cas en cause l'indépendance des assemblées ou le libre choix des collaborateurs. La parole

tendant à réformer les méthodes de travail du Sénat dans le respect du pluralisme, du droit d'amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un Sénat plus présent, plus moderne et plus efficace. Le temps est venu de combler plus efficace. Le temps est venu de combler un vide juridique, afin de contribuer à clarifier le fonctionnement de la vie parlementaire.

Nous avons une bonne occasion de mettre en oeuvre ce précepte. Tout le monde sait ici que s'il n'avait pas été question de Mme Penelope Fillon, personne ne parlerait aujourd'hui des emplois familiaux.

Cet amendement vise à permettre la définition d'un statut des collaborateurs parlementaires répondant aux très nombreuses spécificités de la vie parlementaire, en vue de donner, dans le titre III, un encadrement juridique plus précis à cette profession. L'introduction d'un tel cadre permettrait de lutter efficacement et de manière pérenne contre les emplois appelés « fictifs ».

Il existe une réglementation extrêmement développée, qui fixe des règles de recrutement et de gestion de carrière, avec un salaire minimum, bien au-dessus du SMIC, et une rémunération

le complément salarial d'ancienneté, le complément salarial « jeune enfant », le plan d'épargne entreprise. En outre, des avantages en nature existent : remboursement des frais professionnels, chèques-restaurant, chèques-vacances.

; ce texte le prouve. Ce qui a choqué, dans ces affaires dont on a beaucoup parlé, ce n'est pas tant le fait qu'il s'agissait d'emplois familiaux que le doute sur la réalité de ces emplois et sur le niveau de rémunération associé. Au lieu d'interdire purement et simplement, au lieu d'abattre le troupeau au nom de quelques brebis galeuses, il aurait donc été beaucoup plus logique, beaucoup plus mesuré, beaucoup plus raisonnable, de réglementer davantage cette profession,

pour les élus, qui ne pourront plus embaucher librement, et pour des hommes et des femmes qui, dans leur immense majorité, ont jusqu'à présent fait très correctement leur travail.

pour les membres du Gouvernement. Je rappelle que le décret du 14 juin dernier a fixé la règle de l'interdiction des emplois familiaux pour les cabinets du Président de la République et des ministres.

du Gouvernement. Est également prévue une obligation de remboursement des sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l'interdiction. La commission des lois a modifié l'article 3, avec pour objectif louable de faire respecter le principe de légalité des délits et des peines. Elle a repris la notion de « famille » telle qu'elle est prévue aux articles 4 et 5 pour les parlementaires et les élus locaux. Si, en application de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les crimes et les délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables et la procédure pénale, le principe de séparation des pouvoirs impose au législateur d'assurer une conciliation qui ne soit pas déséquilibrée. C'est ce que propose le Gouvernement par cet amendement, dont la rédaction respecte le principe de légalité des délits et des peines.

qui a jugé possible de renvoyer à une norme inférieure, par délégation de la loi ou du règlement, la définition de certains éléments constitutifs d'une incrimination. Ainsi, la loi peut se borner à fixer le cadre général de la répression, ainsi que les peines applicables, et renvoyer au règlement le soin de préciser le champ d'application et certains éléments de l'infraction. En application de ces jurisprudences, le Gouvernement estime que le pouvoir réglementaire peut parfaitement définir les membres de la famille tombant sous le coup de l'interdiction.

préciser dans quel cas le juge pourra la prononcer. Si la définition de la famille du membre du Gouvernement ne figure pas dans la loi, le juge ne pourra pas

que l'on ne peut pas opposer la séparation des pouvoirs s'agissant de l'application d'un principe constitutionnel de légalité des délits

L'article 3, issu des travaux de la commission des lois, mène à une interprétation inexacte, selon nous, de l'objet de l'obligation d'information. il n'est pas question d'aboutir à l'interdiction des embauches dites « croisées », ce qui serait manifestement disproportionné. Il s'agit de faire en sorte que la HATVP soit informée de l'existence d'un tel lien. L'embauche croisée n'est pas, par par elle-même, constitutive de conflits d'intérêts. En application de l'article 10 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique « lorsqu'elle constate qu'un membre du Gouvernement se trouve en situation de conflit d'intérêts, publique lui enjoint de faire cesser cette situation ». La HATVP n'utilisera ce pouvoir d'injonction que s'il existe une situation de conflit d'intérêts. Il n'est donc pas nécessaire de le préciser dans le projet de loi.

aux membres du Gouvernement qu'aux parlementaires. Cet amendement vise à assurer la publication de la déclaration de parenté concernant un collaborateur ministériel dès lors qu'elle a été enregistrée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Lors de la discussion générale, je vous avais indiqué que le Gouvernement serait prêt à engager des échanges constructifs avec le Sénat sur un certain nombre de sujets.

En effet, comme peuvent en témoigner les nombreux amendements relatifs à la création d'un réel statut, au régime et aux modalités des licenciements, à la portabilité de l'ancienneté à la demande d'un contrôle plus effectif du travail de ses collaborateurs, il s'agit pour vous d'un sujet central. Vous le savez, le projet de loi et le projet de loi organique rétablissant la confiance dans l'action publique ont pour genèse, notamment, des interrogations sur les modalités de recrutement

et de garder en mémoire les interrogations de nos concitoyens sur le rôle des collaborateurs parlementaires. Je sais combien ce rôle est important, vous l'avez tous souligné. Je veux ici rendre hommage au travail de vos assistants, qui ne comptent ni leur temps ni leur énergie pour être présents à vos côtés. Il faut aussi que les Français en prennent conscience. Nos débats peuvent y contribuer.

Le Gouvernement a tout d'abord pris en considération les débats que nous avons eus dans le cadre de la discussion générale. Pour répondre aux attentes exprimées par plusieurs d'entre vous, nous avons décidé de retirer notre amendement tendant à supprimer l'ajout fait par la commission des lois à l'article 6 sur la fin des contrats des collaborateurs. À ce titre, j'exprimerai cependant une une préoccupation du Gouvernement sur les conditions liées au licenciement des collaborateurs parlementaires. C'était le sens de la démarche qui, dans un premier temps, nous avait conduits à déposer cet amendement de suppression.

par des mesures qui ne sont pas comprises par d'autres salariés licenciés, eux aussi se trouvant souvent dans des situations extrêmement difficiles. Je ne méconnais pas les problèmes rencontrés par les collaborateurs parlementaires, en particulier à l'Assemblée nationale, après le fort renouvellement qu'a subi la Chambre. Néanmoins, la situation des collaborateurs parlementaires n'est, me semble-t-il, pas totalement comparable à celle de certaines personnes licenciées pour motif économique,

permettant leur reconversion en assurant une sécurisation financière. Il me semble donc important d'avoir à l'esprit ces éléments, faute de quoi nous pourrions donner collectivement le sentiment de créer à façon un statut spécifique dans un contexte où la plupart des Français ne bénéficient pas de telles dispositions. Sur ce point, et plus largement sur la question des dispositions relatives aux collaborateurs, revendication très ancienne et légitime, le Gouvernement estime qu'il appartient aux assemblées de se concerter pour répondre au mieux, par la voie de la négociation, aux enjeux qui sont posés. Il est important qu'un dialogue se noue. Le Gouvernement est disponible pour y contribuer. Je constate Je constate que de nombreux amendements ont été déposés. Ils expriment votre préoccupation et votre volonté d'améliorer les choses. Je pense en particulier à l'amendement n° 282 de la

Qu'ils soient membres de notre famille ou non, ce sont des collaborateurs engagés qui subissent de très fortes contraintes du fait de notre activité sans horaire et continue durant de longues sessions.

dans les exigences de nos relations avec nos collaborateurs parlementaires. Nous avons avec eux un lien tiré d'un contrat de travail, mais la dispersion de ces collaborateurs dans les bureaux

précisions que je souhaitais apporter au début de cette étape de notre débat, en espérant que nous serons à la fois attentifs à nos collaborateurs et concis dans nos interventions.

L'objet de cet amendement, en coordination avec l'amendement précédent, est de réécrire l'intégralité du titre III du projet de loi rétablissant la confiance dans l'action publique. Il comprend cinq paragraphes pour répondre pleinement à l'exigence de transparence sur l'usage de l'argent public s'agissant de l'emploi des collaborateurs parlementaires. En effet, le présent projet de loi n'aborde la question des collaborateurs parlementaires que par le biais de la suppression de ce qu'il est convenu d'appeler les « emplois familiaux Or, depuis des années, les collaborateurs parlementaires ne bénéficient d'aucun cadre juridique. Cette absence de statut professionnel rend possibles des dérives telles que celles qui ont été révélées à l'occasion, notamment, de l'élection présidentielle. présidentielle. Une telle situation met à mal l'image de l'ensemble des parlementaires et de la profession des collaborateurs parlementaires. Elle a heurté les citoyens soucieux de transparence quant à l'usage de l'argent public mis à disposition des parlementaires dans l'exercice de leur mandat. La moralisation de la vie publique, objet du présent projet de loi, passe donc par la définition d'un statut des collaborateurs parlementaires, inscrivant des règles déontologiques et des garanties sociales répondant aux très nombreuses spécificités de la vie parlementaire. L'amendement

budgétaire mise à disposition, de la nécessité de créer des associations ou du dialogue social. À cet égard, je regrette que, à la suite d'une application quelque peu rigoriste de l'article 40 de la Constitution, une disposition à laquelle nous tenions beaucoup,

n'est pas précisément définie. Cet amendement de repli vise donc à donner une définition précise du métier en précisant que les parlementaires et les groupes parlementaires recrutent librement ces collaborateurs, et que les crédits alloués pour le recrutement servent exclusivement à cet effet.

les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs. Cet amendement prévoit aussi que les parlementaires disposent à cet effet d'un crédit affecté à la rémunération desdits collaborateurs. Le bureau de chaque assemblée, et non le règlement, s'assure de la mise en oeuvre d'un dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.

serviront exclusivement à cet effet, sans aucune autre possibilité. Ce sous-amendement prévoit également de mieux organiser les conditions du dialogue social

parole est à M. Henri Cabanel. Cet amendement a pour objet de réhabiliter le métier de collaborateur parlementaire, à la suite des récents scandales qui l'ont entaché et compte tenu de son opacité aux yeux du grand public. Collaborateur, assistant, attaché ... trois termes pour un point commun : ils maintiennent un contexte flou, alors que les missions font appel à une palette de métiers qu'il faut reconnaître. Il est urgent de jouer la carte de la transparence sur cette profession, dans un double objectif : celui du respect des membres de cabinet parlementaire, dont l'image a été salie, et celui de l'explication de leurs missions auprès des citoyens. Comment jouer cette carte de la transparence ? Par la connaissance de la palette de métiers et d'expertise des membres de cabinet parlementaire et leur reconnaissance. Cet amendement vise à faire en sorte que les membres des cabinets parlementaires soient identifiés à partir de leurs compétences et de leurs missions, comme au sein de toutes les entreprises ou des cabinets de collectivités, de préfectures, de ministères ... Une fiche de poste obligatoire, des entretiens d'évaluation annuels et, surtout, un intitulé de poste sur les missions réelles permettront une clarification des activités.

conformément aux dispositions du code du travail relatives au dialogue social. Ce dialogue social porte, notamment, sur les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité

Le dialogue social porte, notamment, sur les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail. Il détermine la négociation d'accords collectifs.

effet important de mettre en avant la nécessité d'une instance de dialogue social pour les parlementaires employeurs, dès lors qu'il s'agit d'une obligation du code de travail. Notre amendement

causant un tort majeur à nos assemblées, aux parlementaires, à leurs collaborateurs et, plus généralement, à la démocratie représentative. Cet amendement vise donc à doter nos institutions des outils nécessaires pour garantir l'effectivité des emplois de collaborateurs parlementaires et de groupe parlementaire.

D'ici là, et plus généralement, l'inspection du travail et la commission commune aux assemblées et à la Cour des comptes nous apparaissent comme les outils les plus pertinents pour exercer ce contrôle. L'amendement

à l'Assemblée nationale. Près de 1 000 collaborateurs parlementaires ont ainsi été licenciés lors des élections législatives de juin dernier, et un nombre important d'entre eux devraient malheureusement l'être en octobre au Sénat. Sénat. Aux conséquences naturelles des changements de majorité s'ajoutent les conséquences de la fin du cumul des mandats, qui a réduit d'autant les possibilités de reclassement. À la précarité des durées de contrats s'ajoute la précarité des conditions de travail, puisque la moitié des collaborateurs travaille à temps partiel. Si la moyenne des salaires est de 2 800 euros bruts par mois, les disparités sont très importantes entre les collaborateurs, et les mi-temps conduisent souvent à une double activité. Toutes ces raisons ont conduit les syndicats de collaborateurs à demander la mise en place d'une convention collective. Nous soutenons cette revendication. Une

; lorsque nous n'avons plus de mandat, nous sommes une entité qui disparaît, comme n'importe quelle entité qui ne peut plus employer. Il ne s'agit pas pour autant de proposer la création d'un corps de fonctionnaires ! Personne ne l'a demandé.

concitoyens : les parlementaires ne peuvent pas travailler seuls ; celles et ceux qui les accompagnent sont des personnes de qualité qui réalisent un travail remarquable. Il faudra vraisemblablement du temps et de la pédagogie, après ce qui s'est passé pendant la campagne présidentielle, pour rétablir la confiance. Je salue à mon tour la démarche du rapporteur Philippe Bas, qui va nous permettre de réaliser un premier pas,

Nos collaborateurs parlementaires ne sont pas des sous-salariés ; ce sont des salariés à part entière ! Au risque de paraphraser un Président de la République qui distinguait ceux qui ne sont rien de ceux qui réussissent,

le travail de nos collaboratrices et de nos collaborateurs.

ne s'applique pas au Gouvernement. Ainsi, vous pourriez nous aider à mettre en oeuvre l'assimilation

nous proposons une évaluation du travail du cabinet parlementaire par un tiers indépendant, afin de favoriser la transparence de ses activités et de contribuer à la responsabilisation et à la transparence des élus envers les citoyens. Cette évaluation analysera l'adéquation des salaires au temps de travail, à la mission, et elle donnera lieu à la mise en place de, de fiches et d'intitulés de postes, sur le modèle du management des entreprises ou des administrations. Dans le cadre de l'évaluation de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, de mon cabinet parlementaire au mois de septembre dernier, l'évaluateur de l'AFNOR Certification a réalisé pour chaque membre de mon cabinet cette identification des missions, ainsi que les d'organisation et de validation, le tout assorti d'une évaluation du résultat, avec des auditions des parties prenantes- élus, chefs d'entreprise, organismes -, qui a permis de constater l'efficience de notre mode de travail et d'ouvrir des pistes d'amélioration. L'évaluation d'un travail parlementaire, c'est donc possible. C'est d'ailleurs l'une des preuves pour le citoyen que l'emploi n'est pas fictif.

c'est une liberté qu'il a exercée ; ce n'est pas une contrainte qu'il a subie. Chacun d'entre nous peut apprécier les conditions dans lesquelles il souhaite faire évaluer ses collaborateurs sans que lui soit imposée une règle générale. C'est la raison pour laquelle la commission, tout en exprimant sa sympathie pour cette pratique innovante, n'a pas souhaité l'imposer à chacun de nos collègues. L'avis est donc défavorable, mais bienveillant

n° 2 rectifié. Cet amendement prévoit que le bureau de chaque assemblée étudie les modalités de mise en place d'une portabilité de l'ancienneté des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires entre deux contrats et entre les deux assemblées.

enrichissante, mais pour une durée très courte. En parallèle de la valorisation des compétences obtenues et des savoir-faire développés, il est nécessaire d'accompagner la portabilité des droits lorsque des collaborateurs parlementaires deviennent des collaborateurs de groupes parlementaires ou quand ils changent d'assemblée. L'amendement que nous vous proposons va dans ce sens, en retenant l'idée d'une portabilité de l'ancienneté mise en place entre deux contrats et entre les deux assemblées.

portabilité de l'ancienneté, pour reprendre cette expression un peu baroque, mais que chacun peut comprendre, est en partie d'ailleurs satisfaite. En effet, nos

des collaborateurs parlementaires dans les conditions d'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale. Comme l'a précisé ma collègue Brigitte Gonthier-Maurin, avec une durée moyenne de 3,7 ans en poste, les collaborateurs parlementaires ont besoin d'évoluer dans leur carrière : l'accès à la fonction publique territoriale pour des personnes qui se sont investies en faveur de l'intérêt général dans l'institution qui

en séance publique. Nous nous en félicitons. L'idée des syndicats de collaborateurs parlementaires est d'accéder à des passerelles vers la fonction publique territoriale. En effet, si les contrats de travail des collaborateurs parlementaires sont des contrats de droit privé, l'accès aux concours administratifs, y compris la troisième voie, n'est pas une revendication sans intérêt. Alors que l'expérience dans le secteur associatif ou syndical peut être prise en considération dans les années ouvrant la troisième voie, il semblerait logique que l'ancienneté puisse être reconnue pour les collaborateurs parlementaires dans les conditions d'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale. pour présenter l'amendement n° 149 rectifié. Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de notre débat sur la définition des garanties légales que nous pouvons apporter à la profession de collaborateur parlementaire. Il s'agit plus particulièrement ici de parler de leur avenir après le travail parlementaire. Nous proposons d'ouvrir aux assistants parlementaires et aux collaborateurs des groupes politiques du Parlement la possibilité de se présenter aux concours internes de la fonction publique. Actuellement, les assistants parlementaires et les secrétaires des groupes politiques, du fait de la nature de leurs contrats de travail, de droit privé, peuvent se présenter soit aux concours externes de la fonction publique, soit au troisième concours réservé d'ordinaire aux cadres du secteur privé et associatif. Pour information, nous parlons de huit postes en moyenne au cours de ces dix dernières années pour l'École nationale d'administration. Certaines institutions n'ont pas de troisième concours : c'est le cas du Sénat et de l'Assemblée nationale. Sur le fond, il est impossible d'assimiler parfaitement les collaborateurs politiques à des salariés de droit commun. Ces collaborateurs sont rémunérés au moyen de fonds issus de deniers publics. Ils assistent les parlementaires dans l'accomplissement de leurs fonctions de législation, d'évaluation et de contrôle, fonctions qui sont toutes énumérées par la Constitution. Ils concourent, par leur action, à permettre aux élus nationaux de faire vivre le principe, lui aussi constitutionnel, du pluralisme. Enfin, ils sont employés soit directement par des élus, soit par des associations composées exclusivement d'élus, c'est-à-dire des employeurs dont l'activité est exclusive de tout intérêt économique ou commercial. Cette rapide description correspond aux critères traditionnellement retenus par le Conseil d'État pour constater l'existence d'une activité de service public administratif entraînant ainsi, conformément à une jurisprudence constante, l'application aux salariés concernés d'un régime de droit public assimilable à celui d'un fonctionnaire. Une telle reconnaissance contreviendrait bien évidemment à la souplesse nécessaire à l'exercice de fonctions politiques. Pour autant, l'absence de reconnaissance actuelle d'un statut du collaborateur politique ne permet pas de rendre compte des aspects spécifiques de ces emplois et laisse, dans le flou du droit, la porte ouverte aux dérives les plus diverses. Cet amendement offre une solution de compromis permettant à la fois de reconnaître la nature particulière de ces emplois par rapport aux salariés de droit commun, sans pour autant faire des assistants parlementaires et des secrétaires de groupe des fonctionnaires. Il s'agit de leur ouvrir la possibilité de se présenter aux concours internes de la fonction publique, en leur donnant ainsi l'opportunité de reconversion et de valorisation d'un engagement qui, quoique politique, reste fondé sur un attachement certain à l'intérêt général. Je veux remercier ne cessent de me surprendre et de me réjouir : j'ai rarement vu le groupe CRC et le groupe Union Centriste présenter un amendement en tous points identique.

aux concours internes de la fonction publique. Mais les auteurs de ces amendements nous ont rappelé que, même s'il s'agit de contrats de droit privé, il est difficilement contestable que nos collaborateurs concourent

à la fonction publique par la troisième voie ne comporte qu'un nombre de places limitées, je me suis résolu, avec la commission, à émettre un avis favorable sur ces amendements.

mais je vous entends. Comme il s'agit de nouveau de la question des collaborateurs parlementaires, je m'en remets à la sagesse de la

Si les plafonds prévus sont insuffisants, il faudrait les augmenter, plutôt que de passer par des voies détournées. Même si l'on parle d'un épiphénomène, cette mesure sert la transparence ; elle me semble donc de nature à compléter les dispositions proposées par le Gouvernement pour moraliser le recrutement

il semble aujourd'hui que le déficit de publicité autour des offres de recrutement d'agents contractuels fasse obstacle au respect effectif du principe d'égalité d'accès à l'emploi public, et que cette opacité soit de nature à faire naître des doutes sur les critères d'attribution de ces emplois et les risques de népotisme ou d'emplois fléchés.

accessible à tous. Cette mesure présente l'avantage de n'être pas coûteuse, compte tenu de l'existence du site internet de la Bourse interministérielle de l'emploi public, sur lequel certaines offres sont déjà publiées. Il suffit de généraliser cette pratique.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, mon propos est personnel et n'engage en rien mon groupe, pourquoi je ne voterai pas l'article 4, alors même que le projet de loi comporte nombre de dispositions très légitimes et utiles et qu'il part d'une bonne intention. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions ... Ce texte en est par certains côtés une illustration caricaturale. Je prendrai le seul exemple de l'interdiction des emplois dits « familiaux ». Depuis des années, comme cela a été a été souligné à plusieurs reprises, nous critiquons la tentation pour les gouvernements de légiférer à la suite d'un fait divers ou d'un événement marquant, dont on tire aussitôt des conclusions générales. En l'espèce, il s'agit des emplois des membres de la famille Fillon, qui, plus que familiaux, sont surtout des emplois présumés fictifs et rémunérés hors normes. C'est cela qu'il s'agit de prévenir et de sanctionner. familiaux, quitte à créer à l'égard des parlementaires et des membres du Gouvernement une discrimination abusive. Personne

aux politiques une interdiction générale, totalement discriminatoire ? Certes, il est justifié d'attendre des élus un comportement exemplaire et de leur imposer des règles spécifiques, afin d'éliminer, autant que faire se peut, le soupçon. Mais il suffirait pour ce faire d'encadrer strictement les embauches familiales, comme a su le faire le Sénat, en limitant à un seul emploi ce type de recrutement et en plafonnant le niveau de rémunération. La loi pouvait fort bien s'en tenir à cet encadrement, à charge pour chacune des assemblées, si elles sont encore autonomes, d'en préciser les modalités. Or on a choisi la voie de l'interdiction radicale, alors que la notion même de famille, comme on l'a déjà beaucoup souligné, n'a pas cessé de s'élargir et de se diversifier, comme le prouvent d'ailleurs les alinéas de l'article 4 fixant le périmètre de la famille. conduira forcément à mener des investigations sans fin et à encourager la délation, ce qui n'est pas la meilleure potion pour une

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, l'interdiction des emplois familiaux fait suite aux différentes affaires dont nous avons tous été les tristes spectateurs lors de l'élection présidentielle. présidentielle. Il va de soi qu'il est indispensable d'empêcher de telles dérives, car les Français attendent de leurs représentants, au quotidien et en toute circonstance, exemplarité et équité, et qu'ils s'entourent des meilleurs éléments pour les assister dans l'accomplissement de leur mandat de manière efficace. S'il est parfaitement justifié d'encadrer la profession de nos assistants, il faut cependant distinguer l'emploi fictif familial de l'emploi effectif et réel d'un membre de la famille possédant les compétences et les diplômes pour exercer une telle profession.

des règles existent déjà au Sénat en matière de plafonnement du salaire et du nombre d'emplois familiaux autorisés. Il est à mon sens compréhensible qu'un élu puisse être amené à travailler avec une personne compétente qui lui est proche et en qui il a une confiance absolue. Je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que ni ma femme, ni mes enfants, ni un quelconque autre membre de ma famille ne travaillent à mes côtés ou n'aspire à quelque mandat politique que ce soit. Selon moi, les candidats devraient être jugés sur leurs compétences et leurs talents, non sur leurs liens de filiation, quel que soit l'emploi pour lequel ils postulent. Le contraire serait pure et simple discrimination. Je pense à des collaborateurs et collaboratrices parlementaires également « fils ou filles de qui ont accompli un travail remarquable de tous les instants auprès de leur élu et sur lesquels on a jeté l'opprobre de manière éhontée et aveuglément.

d'illégal. Je considère que cette mesure d'interdiction ne saurait à elle seule régler le problème de la moralité inhérente à notre fonction. S'il faut désormais interdire à tout élu de travailler avec un membre de sa famille proche,

La loi pourra, certes, prévoir de longues énumérations de cas d'impossibilité de recrutement, visant notamment les conjoints et enfants, mais elle se révélera impuissante, devant une autre partie, tout aussi importante, mais immergée, du même phénomène, contre laquelle elle risque de n'être que d'une efficacité très limitée. L'amendement

du texte : rétablir la confiance des citoyens dans l'action publique. La priorité est plutôt de s'assurer que les moyens alloués aux parlementaires pour rémunérer leurs collaborateurs soient utilisés à rémunérer des personnes assistant effectivement les parlementaires dans leurs fonctions, au lieu d'introduire des dispositions discriminantes dont les effets sur l'amélioration du travail législatif sont plus qu'hypothétiques. Se tromper de priorité et cibler

d'intégrité, prévenir les conflits d'intérêts et assurer la transparence dans la vie publique. Comme nous le savons, des pratiques récentes ont pu heurter nos concitoyens,

les membres de la famille proche, nous avons évité un cercle trop large. De la sorte, nous ne risquons pas d'enfreindre le droit au respect de la vie privée, non plus que la liberté contractuelle, qui pourrait être invoquée par ailleurs.

Je trouve invraisemblable que l'un d'entre nous ayant un excellent collaborateur, de très grande qualité, qui rencontrerait sa petite-fille- car on va jusqu'aux conjoints de nos petits-enfants

Jean-François Longeot. La suppression des emplois familiaux ne suffit pas à garantir la réalité de l'emploi de certains collaborateurs parlementaires. Le présent amendement tend donc à créer un système de contrôle de l'effectivité du travail des collaborateurs parlementaires. Les récentes affaires impliquant des collaborateurs, également membres de la famille du parlementaire employeur, ont provoqué une forte réprobation parmi les citoyens. Néanmoins, cela a visé en premier lieu non pas la nature familiale de l'emploi,

Cet amendement vise à instituer un contrôle de l'effectivité du travail réalisé par le collaborateur parlementaire dans des conditions fixées par les assemblées. En proposant un contrôle sur la réalité de l'emploi de l'ensemble des collaborateurs parlementaires,

Le scrutin est ouvert.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

Le scrutin est ouvert.